L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d'urgence économiques et sociales

Mme la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, et moi-même tenons, au nom de l'ensemble du Gouvernement, à vous remercier, monsieur le président du Sénat, car, ces jours derniers et dans les délais extrêmement contraints par l'urgence de la situation, vous avez pleinement oeuvré pour créer les conditions propices à un débat de qualité sur le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales. La discussion qui s'engage à présent sous votre présidence intervient quelques heures après le vote de l'Assemblée nationale. Elle approfondira les échanges intenses et précis que nous avons eus mercredi dernier lors de notre audition en commission. Surtout, mesdames, messieurs les sénateurs, cette discussion s'inscrit dans le prolongement du travail étroit que nous avons eu en amont avec les deux chambres grâce notamment à un échange constant entre les rapporteurs Olivier Véran et Jean-Marie Vanlerenberghe. Nous tenons à saluer cette démarche parlementaire à double titre. D'une part, elle témoigne d'un esprit de responsabilité et d'une volonté de participer au rétablissement rapide d'un climat d'apaisement. C'est particulièrement précieux, car, par la désinformation, le rejet de la nuance, la prime au ou au, il n'a jamais été aussi facile d'infuser un climat de défiance, un climat de défiance, de dénigrement de l'autre, d'ironie permanente, parfois de violences, y compris physiques. D'ailleurs, certains élus ont subi des actes d'intimidation, des agressions, que nous devons tous ici unanimement condamner.

Ce lien, vous le savez mieux que quiconque, ne peut exister sans la démocratie, et réciproquement ; c'est un équilibre fragile à maintenir. D'autre part, nous tenons à saluer la démarche parlementaire dans laquelle vous vous inscrivez, car elle participe de notre capacité collective à apporter des réponses à la fois rapides, fortes et concrètes pour nos concitoyens afin que chacun puisse vivre décemment de son travail et choisir sa vie professionnelle. cette capacité collective à concrétiser une société de l'émancipation par le travail et la formation, rompant avec les droits formels et avec le déterminisme de naissance ou géographique, qui est fortement questionnée aujourd'hui. aujourd'hui. Pour réaliser ce projet de société, le Gouvernement a engagé depuis dix-huit mois une profonde transformation de notre modèle économique et social, conformément aux engagements pris par le Président de la République devant les Français.

est le sens du dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, de la complémentaire santé pour des soins de bonne qualité au prix de 1 euro par jour ou de la prise en charge progressive de 100 % des frais de soins dentaires, d'optique ou de prothèses auditives. aussi le sens de l'action menée en matière d'apprentissage, de formation professionnelle, ainsi que de développement et d'attractivité du territoire. Voici notre cap : stimuler la croissance et la rendre riche en emplois et inclusive.

Certains de nos concitoyens n'ont pas ce temps, car leur horizon, alors même qu'ils travaillent ou ont travaillé toute leur vie, n'est pas la fin du mois, mais le 20, voire le 15 du mois. Comment, dans ces conditions, ne pas s'inquiéter pour ses enfants, ses petits-enfants ? Comment se projeter dans l'avenir ? Pour citer André Gide, certains de nos concitoyens éprouvent le sentiment que « le présent serait plein de tous les avenirs, si le passé n'y projetait déjà une histoire En clair, beaucoup de nos concitoyens désespèrent de ne plus pouvoir espérer ! Ce désespoir de vies empêchées, cette souffrance, cette colère se sont exprimés très fortement depuis plus d'un mois, matérialisés par le mouvement des « gilets jaunes ». Cette colère, cette souffrance nous interrogent collectivement sur notre capacité à apporter des réponses de long terme, qui transformeront la situation, mais en même temps des réponses qui soient rapides, Apporter des réponses rapides, c'est la condition de l'apaisement. C'est l'objet de l'état d'urgence économique et social qui a été décrété par le Président de la République le 10 décembre dernier. Le présent projet de loi en est la traduction. Comme vous le savez, il contient quatre mesures fortes.

la CRDS. Bien évidemment, elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime d'activité. La deuxième mesure concerne les heures supplémentaires : elle permet à tous les salariés et les fonctionnaires qui réalisent des heures supplémentaires, soit environ 9 millions de personnes de ne payer désormais ni cotisations salariales ni impôt sur le revenu, à concurrence d'une rémunération annuelle nette au titre des heures supplémentaires de 5 000 euros. Si vous la votez, cette mesure entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2019.

même si, il faut le rappeler, 40 %, les plus modestes, en avaient été exonérés d'emblée. Le projet de loi rétablit, à compter du 1 janvier 2019, le taux de CSG de 6,6 % pour la moitié des retraités qui avaient supporté la hausse de 1,7 Ce sont 3,8 millions de foyers, 5 millions de retraités, qui vont bénéficier de ces dispositions. Concrètement, pour un retraité percevant une retraite, avant cotisations sociales, de 1 600 euros et sans autre revenu par ailleurs, ce sera un gain de pouvoir d'achat de 325 euros sur l'année. Avec cette mesure, seuls 30 % des foyers fiscaux avec un retraité auront un taux de CSG de 8,3 % et 70 % ne seront plus touchés par la hausse.

la prime d'activité allie deux impératifs : le travail, qui doit mieux payer, et la justice sociale. Grâce au choix que nous faisons d'un renforcement de la prime d'activité, 100 % des personnes qui n'ont que le SMIC pour vivre auront bien 100 euros nets par mois de revenus supplémentaires dès 2019, 100 % des personnes seules- femmes ou hommes -avec enfants qui n'ont pour vivre qu'un salaire n'excédant pas 2 000 euros par mois auront bien 100 euros de plus et

et le jour même de sa transmission au Sénat par l'Assemblée nationale. Il faut l'admettre, ce sont des conditions de travail peu confortables. Heureusement, ce projet de loi est court : il ne compte que quatre articles, eux-mêmes relativement brefs. En outre, je tiens à souligner la bonne collaboration des services du Gouvernement, qui ont répondu avec rapidité et précision à nos questions. Je les en remercie vivement. Le dialogue a également été nourri ces derniers jours avec le rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale, Olivier Véran, dont je salue ici la disponibilité, l'esprit d'ouverture et la courtoisie.

est qu'on ne les écoute pas. Nous pouvons souvent dire au Gouvernement qu'il ne nous entend pas. Nous n'en serions sans doute pas là s'il avait suivi le Sénat sur la CSG et sur le gel des taxes sur le carburant. Ce n'est Ce n'est pas un reproche personnel, mesdames les ministres, monsieur le ministre. Il s'adresse de manière générale à tous les gouvernements depuis des décennies. Venons-en au fond des mesures de ce projet de loi. Il s'agit, comme vous le savez, mes chers collègues, de traduire en droit les mesures annoncées par le Président de la République.

Précisons qu'il s'agit des employeurs soumis à l'obligation de contribuer à l'assurance chômage et de certains autres employeurs à statut particulier, mais pas de la fonction publique.

il faut avoir de la patience ... J'en ai pour l'éternité ! En revanche, les cotisations patronales ne seront pas exonérées. Il n'y a donc pas d'incitation, maintenant vers la gauche de notre hémicycle -, à privilégier l'usage d'heures supplémentaires par rapport à l'embauche de nouveaux salariés. C'est simplement une mesure de pouvoir d'achat renforcé pour les salariés. L'article 3 rétablit un taux de CSG de 6,6 %, c'est-à-dire le taux applicable jusqu'en 2017, sur les pensions de retraite et certains revenus de remplacement pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain seuil. Ce seuil correspond à un revenu net mensuel de 2 000 euros pour une personne seule et de 3 060 euros pour un couple. Enfin, l'article 4 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement six mois après la promulgation de cette loi afin de dresser le bilan de la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité prévue le 1 janvier prochain. Une fois n'est pas coutume, une telle demande de rapport est opportune. D'abord, parce qu'elle nous permet de débattre aujourd'hui dans cet hémicycle de la prime d'activité. Ensuite, parce que, pour cette mesure, plus encore peut-être que pour les autres, l'application concrète de la loi sera capitale.

droit. Mesdames les ministres, le rapport du Gouvernement devra être précis sur ce point ; il devra présenter des pistes pour améliorer, si nécessaire, ce taux de recours. L'Assemblée nationale a adopté quelques amendements Il s'agissait essentiellement d'apporter certaines précisions, souvent utiles d'ailleurs. Pour autant, aucun d'entre eux n'a modifié l'économie générale du texte. Les mesures de ce projet de loi sont donc substantielles. De plus, elles s'inscrivent dans un plan plus vaste comprenant en particulier l'abandon des augmentations

Par conséquent, d'un point de vue juridique, tout ce que le Parlement votera devra être compensé à la sécurité sociale, sauf à ce qu'une loi de financement de la sécurité sociale prévoie le contraire. À titre informatif, vous trouverez, dans le rapport de la commission, les tableaux d'équilibre pour 2019 rectifiés, si d'aventure le Gouvernement était tenté d'appliquer les principes qu'il a définis dans son rapport de juillet 2018 sur la rénovation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale et que l'on peut résumer par la formule : « que chacun finance ses pertes » ! Les régimes obligatoires de base et le FSV afficheraient un déficit consolidé de 2,8 milliards Nous serions donc assez loin du retour à l'équilibre annoncé au début de l'automne. Comment mieux illustrer la pertinence de nos réserves sur les coupes prévues dans le flux de TVA à à destination de la sécurité sociale et sur le fait que l'on ne saurait lui « faire les poches » avant qu'elles ne soient pleines ? Sous le bénéfice de ces observations, la commission a considéré que l'économie générale de ce projet de loi répond, au moins en partie, à plusieurs préoccupations soulevées par le Sénat, notamment lors de l'examen des deux derniers qu'entraîneront ces mesures, en particulier pour les travailleurs et les retraités aux revenus modestes, seront substantiels. De plus, la commission a considéré qu'il était nécessaire que les propositions faites par le Gouvernement en réponse aux annonces du Président de la République puissent rapidement rapidement se traduire dans les faits. C'est pourquoi elle a adopté le texte transmis par l'Assemblée nationale sans modification et préconise son adoption conforme par le Sénat. est à M. le président de la commission.

à opposer l'exception d'irrecevabilité que nous présentons est spontanée. Elle est le fruit d'une grande incompréhension et, je dois le dire, d'une grande colère. Cette motion, qui soulève l'inconstitutionnalité, vise le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales qui nous est soumis dans la plus grande précipitation. que les conditions de débat, en particulier la grave mise en cause du droit d'amendement, portent un sérieux coup à ce projet dont les conditions d'élaboration ne respecteront donc pas la Constitution. Avant d'en venir aux éléments juridiques précis qui fondent notre motion, je voudrais rappeler d'un mot le contexte social du débat en cours, sur lequel mon amie Laurence Cohen reviendra plus précisément dans le cadre de la discussion générale. Nous assistons à une révolution citoyenne d'ampleur, à un mouvement social inédit, massivement soutenu par la population aujourd'hui encore, malgré toutes les tentatives de dénigrement. Ce mouvement bouscule profondément les dogmes libéraux qui encadrent les politiques gouvernementales depuis vingt ans. Ce mouvement porte sur le pouvoir d'achat, sur la justice fiscale, bien sûr, et nous reviendrons fortement sur ces aspects dans le débat, mais il porte en lui une aspiration formidable à la participation des citoyens non seulement au débat, mais aussi à la prise de décisions. Le peuple n'en peut plus de ces institutions qui autorisent le reniement des engagements et tiennent éloignés de manière de plus en plus évidente les citoyens des élus, en particulier nationaux, sans évoquer le Président de la République, enfermé aujourd'hui dans une posture jupitérienne. Nous n'avons pas attendu aujourd'hui, avec beaucoup d'autres, pour souligner la crise politique et institutionnelle profonde que traverse notre pays. L'abstention croissante aux différentes élections en est un symptôme frappant. Nous constatons, avec cette entrée en force des « gilets jaunes » dans le paysage politique et social, car c'est un mouvement politique et social, que le peuple tente de reprendre en main la situation en rappelant avec force cette volonté de vivre dignement, ce ras-le-bol de l'exposition indécente des richesses en croissance infinie, cette volonté de démocratie. Cette volonté de prendre la parole, de reprendre le pouvoir s'exprime avec l'exigence du référendum d'initiative populaire plébiscité- vous devez entendre cela au Gouvernement et dans la majorité des assemblées -par 78 % des femmes et des hommes de notre pays. Emmanuel Macron, pris de court, a présenté ses propositions à la source du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Outre le fait que ces mesures sont notoirement insuffisantes et relèvent, pour l'essentiel, d'une véritable manipulation des chiffres, tout le monde a été frappé par l'absence de planification en matière de financement et chacun a relevé que les riches étaient protégés de tout effort de participation réelle, pérenne à l'effort de solidarité nationale. La question du financement de votre projet est au coeur du débat. Il est un élément clef de la discussion. Ne pas le reconnaître relève, il faut le dire, d'une forme de malhonnêteté intellectuelle. ? La collectivité, y compris ceux qui bénéficieront de ces quelques miettes, ou bien les détenteurs des plus gros patrimoines, ceux qui profitent du fruit du travail de ces femmes et de ces hommes en lutte, les actionnaires en un mot ? Les plus riches participeront-ils à cet effort d'aujourd'hui et celui, nécessaire, à venir ? Nous avons déposé des amendements importants liés directement, intimement à ce texte, car ils concernent son financement. Ils portent, par exemple, sur la mise à contribution de l'ISF, sur la mise à contribution d'une taxe spécifiquement prévue à cet effet ou sur la mise à contribution de la remise en cause des mesures se substituant, dans la dernière loi de finances, au CICE, cette manne de cadeaux aux entreprises, les plus grandes en particulier, sans contrepartie. Ces amendements, la majorité sénatoriale, sous le regard bienveillant et redevable du Gouvernement et d'Emmanuel Macron, les déclarera sans doute irrecevables. Le principe de cette irrecevabilité a d'ailleurs été décidé avant même le dépôt de nos amendements, puisque le président de la commission des affaires sociales a clairement affirmé ce matin, lors de la réunion de la commission des affaires sociales, que tout amendement ne portant pas sur le corps du texte serait refusé pour des raisons d'urgence. Monsieur le président du Sénat, cette urgence, cette efficacité, c'est précisément cela qui vous avait fait entrer dans une forme de résistance au projet de loi de révision constitutionnelle portée par le chef de l'État. Vous avez, avec le président de la commission des lois, avec la majorité sénatoriale, en vous appuyant sur les groupes d'opposition, mis en avant la défense du droit d'amendement. Vous savez très bien que l'article 3 du projet de loi, entre autres dispositions, limitait fortement le droit fondamental en modifiant l'article 41 de la Constitution. Cet article 3 instaurait l'irrecevabilité de tout amendement sans lien direct avec le projet ou la proposition de loi en discussion. C'est la règle ! Il y a une contradiction manifeste entre l'attitude de votre majorité à l'encontre du projet de loi constitutionnelle et le fait que vous permettiez l'adoption conforme d'un texte qui ne met en cause ni le patronat ni les plus riches. Mais, surtout, quelle profonde incompréhension du mouvement en cours et à la formidable aspiration au débat, à la concrétisation pleine et entière de la citoyenneté ! Le Gouvernement prône un grand débat, mais ce débat est tué dans l'oeuf au Sénat par une lecture tronquée de la Constitution, par une interprétation abusive de ce texte très imparfait, mais qui préserverait quelque peu, du fait de la tutelle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur l'ensemble de nos institutions, le droit d'amendement. La révision de 2008 précisé explicitement la force du droit d'amendement en substituant, à la demande du Sénat et de son rapporteur, Jean-Jacques Hyest, à la notion de limite au droit d'amendement

étions là ! ... le concept de conditions pour exercer le droit d'amendement rappelé dans l'article 44 de la Constitution. L'article 45 rappelle, quant à lui, la possibilité, en première lecture, de déposer des amendements ayant un lien, certes, mais même indirect- j'insiste sur ces termes -, avec le texte en discussion. Sur le site internet du Sénat, rappel de l'alinéa 1de l'article 45 de la Constitution au sujet des cavaliers législatifs : « Tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. » Le site précise aussi que, pour apprécier l'existence d'un lien direct ou indirect, il convient, comme l'a fait le Conseil constitutionnel, de recourir à la technique du faisceau d'indices. Les indices ou les références sont au nombre de trois : l'intitulé, l'exposé des motifs et l'objet du texte. Mesdames les ministres, monsieur le président de la commission des affaires sociales, pouvez-vous maintenir que proposer de débattre des modalités de financement, sans créer de dépenses supplémentaires, bien entendu pour respecter l'article 40 de la Constitution que nous combattons par ailleurs, n'a pas de lien indirect et ne répond pas au faisceau d'indices évoqués ? Tout cela n'est pas sérieux Nous assistons à un coup de force. Nous ne pouvons croire que « la trêve des confiseurs » serait la justification d'une violation de la Constitution. Vous ne voulez, ni au Gouvernement ni à la droite de l'hémicycle, de ce débat, car il touche au fondement de votre politique : imposer, maintenir coûte que coûte l'injustice fiscale et sociale. Vous concédez quelques mesurettes qui, pour ceux qui n'ont rien, apporteraient évidemment un très maigre réconfort pour mieux préserver l'austérité. Solennellement, je vous appelle, en cette fin de journée, à la responsabilité. Un vent se lève dans notre pays, et ne croyez pas qu'il va perdre de sa force dans les jours à venir. Votre responsabilité, notre responsabilité est grande pour ouvrir nos institutions au débat, aux citoyens, pour répondre à cette attente formidable. Si vous décevez cette attente par des mesures de cadenassage comme aujourd'hui, vous devrez répondre demain d'un discrédit définitif de notre Parlement. Monsieur le président du Sénat, levez les irrecevabilités décidées, il y va de la crédibilité et de la dignité de notre assemblée ! Y a-t-il

mais, quand il y a urgence, quand des décisions doivent être appliquées au 1 janvier, personne en France ne comprendrait que le Parlement bloque, personne en France ne comprendrait que nous fassions de la politique politicienne pour empêcher ces mesures de s'appliquer. Ce n'est pas le sujet ! Nous pourrons discuter lors du collectif budgétaire. Nous-mêmes, nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout,

on l'a vu et on le constatera, ne font pas le compte par rapport aux attentes. Voilà la problématique ! Notre motion d'irrecevabilité est un geste fort pour dire au Gouvernement que les parlementaires ne sont pas aux ordres

avait appelé à une application plus stricte des irrecevabilités constitutionnelles, ce qui n'exclut pas de faire

Ainsi que l'a d'emblée annoncé le président Gérard Larcher, le Sénat devrait adopter le projet de loi qui nous est soumis, comme l'a adopté, ce matin, la commission des affaires sociales. Nous avons la volonté, très ferme et très claire, de l'apaisement. Ces dernières semaines ont été difficiles et, dans ce déferlement de colère qui a secoué le pays, n'en déplaise aux apôtres de la violence politique, je lis plus d'autodestruction que d'élan créateur. Eh oui, malheureusement ! La France, que nos voisins jugent arrogante et moquent gentiment comme la « grande nation », est rongée par le doute et, pour emprunter le mot du poète Pessoa, par « l'intranquillité ». Tout à fait ! L'élan collectif semble brisé, la fierté d'un certain modèle, envolée, la possibilité d'un avenir meilleur, évanouie. Nous connaissons bien, tous, ce paradoxe qui fait voisiner dans notre pays une relative satisfaction individuelle et la déprime collective. Nous l'entendons souvent, cette idée que le pays se perd, que la situation ne pourrait être pire, qu'il faudrait alors précipiter les choses et tout jeter aux orties. cela, dont rien n'est, malheureusement, très nouveau, s'exprime souvent dans nos départements. Quelque chose, pourtant, s'est déclenché ces dernières semaines. Tout en étant humble dans les explications avancées, tant le mouvement à l'origine de nos travaux est hétérogène et composite, je voudrais évoquer trois éléments. Le premier, c'est l'extrême sensibilité fiscale à laquelle nous sommes parvenus : le poids des prélèvements et leur raffinement de complexité alimentent la méfiance et le sentiment d'injustice. Dans ce contexte, le bouleversement auquel s'est livré le Gouvernement avec l'augmentation de la CSG a nourri une exaspération bien présente. Le deuxième élément, c'est la délicate promesse, associée à ces changements fiscaux, du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat dépend, vous le savez, de multiples facteurs : la durée du travail, la taille de la famille ou encore le lieu d'habitation. Durant la période récente, nous savons par exemple que le pouvoir d'achat a augmenté, mais, la taille des familles ayant diminué, cette augmentation ne se traduit pas concrètement pour tous. Le pouvoir d'achat- faut-il le rappeler ? -dépend avant tout de l'emploi et l'emploi de la croissance, qui nous fait si cruellement défaut depuis dix ans. Au vu de l'état de nos finances publiques, le pouvoir d'achat distribué par l'État, ce sont, mes chers collègues, des impôts ou de la dette, c'est-à-dire, à terme, la même chose. Avoir mis le doigt dans cet engrenage par des promesses inconsidérées était donc, pour le Gouvernement, à tout le moins hasardeux et le restera, sans doute, encore plus dans

troisième élément que je voudrais souligner, c'est le style et certains propos de l'exécutif, dont les effets ravageurs ont été sous-estimés, mais que nous payons aujourd'hui au prix fort. René Char, poète qui m'est cher, évoquait « l'hémophilie politique de gens qui se pensent émancipés. Combien sont épris de l'humanité et non de l'homme ! Pour élever la première, ils abaissent le second ». Certains de nos concitoyens se sont sentis abaissés, et ce sentiment, bien plus que l'insuffisance de revenus, est difficile à réparer. Alors, oui, nous voterons ce texte s'il peut contribuer à l'apaisement, sans enthousiasme cependant. Certes, les mesures que le Gouvernement propose- la défiscalisation des heures supplémentaires, la CSG des retraités -ont, pour certaines, été proposées, voire adoptées par notre assemblée, mais elles l'ont été dans le cadre cohérent des textes financiers, avec le souci d'en respecter les équilibres et la vision d'ensemble. Le Parlement vient de voter un projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont l'équilibre proclamé était inédit depuis deux décennies. À la différence de ce que vous avez dit en commission des affaires sociales, mesdames les ministres, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un débat technocratique. Ce que l'on appelle familièrement le « trou de la sécu » parle à nos concitoyens. Le fait que, depuis vingt ans, en dépit des hausses d'impôt et de cotisations, notamment de retraite, l'équilibre ne soit pas atteint alimente la méfiance et la crise de confiance dans l'action publique. C'est pourquoi la commission des affaires sociales s'est élevée contre la ponction anticipée des excédents à venir de la sécurité sociale et c'est pourquoi elle demande que la règle de compensation s'applique aux mesures que l'on pourrait qualifier de nouvelles niches fiscales et sociales qui nous sont proposées. Je rappelle au passage que les exonérations de TEPA étaient compensées. La commission s'est également opposée à la sous-indexation des prestations sociales, mesure de bouclage budgétaire, qui est pour nous un dysfonctionnement. Nous aurions souhaité être entendus. Les annonces présidentielles ont été entourées d'une certaine confusion. Tout en comprenant le choix de la prime d'activité dans un contexte où la lutte contre le chômage, lequel est encore beaucoup trop élevé, doit rester notre premier combat et où les entreprises n'ont pas restauré leur situation financière d'avant la crise, les annonces de montants nets risquent de susciter bien des déceptions. Alors, oui, nous adopterons ce projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales. Avons-nous, mes chers collègues, réellement le choix après ce qui vient de se passer ? étant, à nos concitoyens, à nos mandants, nous devons non seulement l'écoute et l'empathie, mais aussi le respect et la vérité. La confiance dans l'avenir ne viendra pas de ce panier de mesures, mais de l'investissement dans la santé, l'éducation et la formation, conditions de l'émancipation sociale.

en 1985, il y a plus de trente-quatre ans, Coluche lançait les Restos du coeur pour apporter aux personnes démunies des repas gratuits. En 1995, il y a plus de vingt-quatre ans, le candidat à la présidence de la République, M. Jacques Chirac, nous parlait de la fracture sociale de notre société. Aujourd'hui, des hommes et des femmes démunies, victimes de cette fracture sociale, se mobilisent. Des Françaises et des Français, des femmes et des hommes en colère, en souffrance, revêtent une chasuble haute visibilité pour être vus, mais, surtout, pour être entendus. Ce mouvement regroupe des milliers de travailleurs et de retraités, modestes, qui ne s'y retrouvent plus. Ce sont les « gilets jaunes ». Des décennies de politiques ont cherché à soigner. Elles n'ont pas guéri pour autant. Aujourd'hui, les plaies sont béantes. Il nous appartient de les soigner. À cet égard, il n'est plus l'heure de se rejeter la faute. Il n'est plus l'heure de se dédouaner sur tel ou tel parti, sur tel ou tel gouvernement. Les « gilets jaunes » méritent mieux. L'heure est venue d'assumer, d'assumer en dépassant toutes les sensibilités politiques, quelles qu'elles soient. L'heure est venue de reconnaître que le désespoir et la détresse de ces Français modestes ne datent pas d'aujourd'hui, ni d'hier, mais d'avant-hier, et que tous les gouvernements, le nôtre y compris, qui se sont succédé ces quarante dernières années n'y ont pas fait suffisamment face. Aujourd'hui, mes chers collègues, le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales, que nous nous apprêtons à examiner, apporte des réponses concrètes, visibles, à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Il s'agit là de premières réponses. Elles devront être suivies par d'autres, en particulier grâce au grand débat national qui sera lancé en janvier 2019.

Il nous appartient d'apaiser pour mieux soigner. Il nous appartient d'apaiser pour mieux panser. Si nous échouons, nous ne pourrons éloigner le tumulte et la fureur qui ont vu le jour en marge de ce mouvement et qui s'échinent à le disloquer et à le dévoyer.

prime sera augmentée pour les travailleurs les plus modestes. À ce titre, l'État assume pleinement son rôle social, en choisissant d'instaurer une hausse immédiate de 90 euros au travers de la revalorisation réglementaire de la prime d'activité. En tenant compte de la hausse du SMIC, nous arrivons à 100 euros nets. Concrètement, grâce à cette mesure, le nombre de foyers pouvant bénéficier de la prime d'activité passera de 3,8 millions à 5 millions, et ce dès le 5 février 2019.

En procédant ainsi, le Gouvernement ne cible pas seulement les bénéficiaires du SMIC : il répond à un panel beaucoup plus large de personnes modestes. Il s'agit bien là d'une réponse sociale et éthique donnée aux travailleurs les plus modestes. Elle doit engendrer la confiance. la seconde mesure sociale. L'effort que nous avions demandé aux retraités par le biais de la CSG était trop important. Ah ! Nous nous sommes trompés, nous l'assumons. « J'assume », permet un retour au taux de 6,6 % jusqu'à 2 000 euros nets de pension pour un retraité célibataire. Ainsi, 70 % des foyers de retraités ne seront plus concernés par le taux maximal de la CSG. Les deux autres mesures répondent à une urgence économique. À cet égard, il est essentiel que l'entreprise prenne, elle aussi, sa part de responsabilité. Durant les dix-huit derniers mois, nous avons permis aux entreprises de se stabiliser, de reconstituer leurs marges et de redevenir compétitives sur la scène internationale. Elles ont sauvegardé les emplois, réinvesti mais les embauches balbutient et les augmentations de salaire tardent. À l'évidence, le mouvement est lent et ne répond pas à l'urgence sociale du moment : on constate un vrai décalage. Cependant, nous demeurons convaincus qu'une nation ayant un tissu d'entreprises qui se porte bien permet à tous de mieux vivre ensemble.

Plus concrètement, cet article prévoit le versement d'une prime de fin d'année pouvant aller jusqu'à 1 000 euros, pour les salariés gagnant jusqu'à 3 600 euros par mois, sans charges ni impôt est inédit. En outre, par son article 2, le projet de loi exonère de charges salariales et d'imposition sur le revenu les heures supplémentaires, plafonnées à 5 000 euros nets par an. Le gain de pouvoir d'achat sera d'environ 500 euros nets pour une personne rémunérée 1 500 euros nets et faisant deux heures supplémentaires par semaine. Mes chers collègues, ce projet de loi permet aujourd'hui à l'État de remplir son rôle social, en redonnant aux travailleurs et aux retraités modestes la capacité d'aller de l'avant de ses articles 3 et 4. Dans le même temps, le Gouvernement aurait pu renoncer à ses promesses qui permettent aux entreprises de retrouver le chemin de la croissance, en supprimant provisoirement la bascule du CICE vers la réduction des charges. Dès lors, le déficit de l'État aurait été bien en deçà des 3 %.

Ce sont les entreprises, et elles seules, qui sont en capacité de définir la juste rémunération du travail et de relancer, avec nous, l'ascenseur social. C'est pourquoi, dans cette confiance renouvelée, nous voterons ce projet de loi sans modification.

Cohen. Monsieur le président, mesdames, monsieur les ministres, mes chers collègues, lors de son allocution du 16 octobre dernier, le Président de la République avait annoncé qu'il refusait de se soumettre et de changer de politique. deux mois plus tard, et après une très large mobilisation populaire dans l'ensemble du pays, M. Emmanuel Macron a dû, pour la première fois depuis son élection, reculer sur les mesures fiscales de taxation de l'énergie

fédérer les luttes. Il a démontré qu'il était possible d'ouvrir une brèche dans la politique jupitérienne. On aurait pu espérer que le Gouvernement sorte davantage et plus tôt de sa bulle dorée pour se rendre compte de la réalité du sentiment d'injustice, qui, à juste titre, traverse notre pays. Malheureusement, il n'en est rien. Le cahier de doléances des « gilets jaunes » était pourtant très clairement articulé autour de mesures en faveur du pouvoir d'achat- hausse des salaires, SMIC à 1 300 euros nets par mois, augmentation des pensions de retraite -et de mesures en faveur de la justice fiscale, en particulier le rétablissement de l'ISF pour faire en sorte « que les gros payent gros et que les petits payent petit ». M. Macron, le président de la finance, a refusé de revenir sur sa politique de cadeaux fiscaux sans contrepartie aux plus fortunés et aux grosses entreprises. Il a maintenu la et la suppression de l'ISF, alors que la majorité des Françaises et des Français y est ministres, les injustices sont flagrantes dans notre pays et elles ne sont plus supportables. Il n'est plus supportable que le PDG de LVMH gagne en une journée ce qu'un salarié moyen de son entreprise gagne en plus d'un an ou que le PDG de Carrefour gagne 553 fois le SMIC. Les richesses produites dans notre pays sont gigantesques. Pourtant, elles ne profitent qu'à une extrême minorité : les actionnaires du CAC 40. Le Gouvernement a refusé de s'y attaquer. Il a préféré les pseudo-solutions que sont la défiscalisation des heures supplémentaires, la fausse hausse du SMIC, financée par les contribuables, la prime exceptionnelle sans impôt ni contribution

; et la prise de conscience de M. Macron est restée bien relative, puisque la hausse de la CSG est simplement annulée pour une partie des retraités, et uniquement pour 2019 pour 2019 ! La droite sénatoriale avait fait voter le recul de l'âge de départ à la retraite pour compenser cette hausse. Notre groupe, lui, s'y était opposé. Il avait fait d'autres propositions de financement, notamment en mettant à contribution les revenus financiers des grandes entreprises.

pour accomplir diverses démarches et réactualiser sa situation tous les trois mois ! Enfin, cette prime est limitée, puisqu'elle ne concernera pas les fonctionnaires. Or 40 % d'agents publics sont au niveau du SMIC ; dans la fonction publique territoriale, les 75 %. La défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires, présentées comme un gain annuel de 155 euros, constituent, elles aussi, un leurre. En réalité, en incitant les salariées et les salariés à effectuer plus d'heures supplémentaires, l'on provoquera une augmentation de la durée du temps de travail au détriment de l'emploi.

comment cette mesure va-t-elle bénéficier aux personnels soignants et non soignants des hôpitaux et des EHPAD, alors qu'ils voient leurs heures supplémentaires exploser sans contrepartie financière et sans possibilité de récupération ?

« En utilisant le budget de la sécurité sociale pour réduire le déficit de l'État, votre gouvernement se livre au plus grand hold-up du siècle. » Vous pourrez utiliser à loisir les ressources de la sécurité sociale, payées par les assurés sociaux, pour renflouer les caisses de l'État. regrettable que la prime exceptionnelle ne soit pas une obligation pour les grandes entreprises qui réalisent des profits colossaux. Mesdames, monsieur les ministres, ces mesures ne font pas le compte. Les femmes en sont particulièrement exclues ; or elles sont souvent parmi les plus précaires. Les Françaises et les Français ne sont pas dupes. Malgré l'écran de fumée que vous répandez afin de masquer vos choix profondément inégalitaires, ils voient bien que les plus fortunés ont droit à toutes vos largesses. Vos largesses, ce sont 40 milliards d'euros pour les grandes entreprises et les actionnaires, sans aucune contrepartie, contrepartie, le remboursement du CICE pour l'année 2018 et la baisse des cotisations patronales, voire leur suppression, décidée pour 2019 ; il s'agit là d'une mesure inique adoptée, ici même, avec la droite sénatoriale. Vos largesses, c'est aussi le maintien de la suppression de l'ISF, soit 4,2 milliards d'euros offerts au détriment d'une politique de justice sociale pour toutes et tous. D'un côté, de somptueux cadeaux de Noël ; de l'autre, des miettes : mais la brèche est ouverte, car vous venez de démontrer que la sacro-sainte loi des 3 % de déficit du pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne n'est pas indépassable. La prise de conscience gagne du terrain : c'est une bonne nouvelle, et vos premiers reculs en appellent d'autres. L'argent existe pour répondre aux besoins des populations, non pour être détourné vers la finance, au détriment de l'humain

Monsieur le président, mesdames, monsieur les ministres, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, « les pays développés dont l'impôt sur le revenu des personnes physiques est relativement peu progressif ont peut-être la possibilité de relever les taux marginaux d'imposition supérieurs sans entraver la croissance économique. Différents types d'impôts sur la fortune peuvent aussi être envisagés

Nous le savons tous ; en mesurons-nous vraiment les conséquences ? La mondialisation, le dogme de la concurrence qui tue la notion de service public, l'évolution du capitalisme au seul service des actionnaires, en creusant partout les inégalités, en ne permettant plus de vivre dignement du fruit de son travail, ont alimenté une bombe qui vient d'exploser chez nous. Ces déflagrations remettent en cause notre fonctionnement démocratique, valident la violence comme moyen d'obtenir des résultats et affaiblissent encore un peu plus- comme si c'était nécessaire -les corps intermédiaires. chers collègues, la grille de lecture de l'action publique doit placer au premier plan l'objectif de lutte contre les inégalités sociales, l'objectif de justice fiscale. En effet, cette dernière conditionne l'acceptabilité de l'impôt, qui permet la redistribution.

relevant de ce projet de loi, et par une quatrième, l'extension de la prime d'activité. L'axiome étant posé de la non-majoration du SMIC au-delà de 1,5 %, ces mesures, qui corrigent des décisions antérieures, permettront des améliorations du pouvoir d'achat.

Pourquoi avoir ignoré, en début de révolte sociale, la proposition constructive du leader d'une centrale syndicale ? En outre, vous ne revenez pas sur certains choix qui porteront atteinte à l'élaboration d'une société solidaire ; je pense en particulier à la désindexation des retraites, pensions et prestations familiales. sur un coût estimé à 10 milliards d'euros pour l'ensemble des dispositifs, 6 milliards d'euros viendront augmenter le déficit budgétaire et la dette. Parce que l'objectif, auquel on peut souscrire, de renforcer la compétitivité de nos entreprises conduit à l'absurdité de doubler le CICE en 2019, parce que le Gouvernement s'entête dans la non-contribution à l'effort des plus aisés de notre pays, vous vous heurterez, mesdames, monsieur les ministres, à une équation impossible. Dans un contexte européen où le besoin d'autorité l'emporte sur celui de liberté, les fondements de notre vivre ensemble et de notre démocratie pourraient en être gravement ébranlés. Très bien

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, dans quelques heures sans doute devrait s'achever le premier chapitre d'une séquence inédite, et qui fera assurément Nos concitoyens l'attendent évidemment avec impatience, ce qui rend notre responsabilité d'autant plus importante. Cette séquence est inédite par l'ampleur de la mobilisation sociale qui a parcouru le pays ; inédite par la colère qui s'est exprimée bien au-delà de la seule question de la fiscalité des carburants aussi, par le désespoir ressenti face aux inégalités qui persistent dans tous les territoires ; inédite par la violence, inacceptable, qui s'est également manifestée, et que nos forces de l'ordre ont su contenir avec professionnalisme et avec leur sens du devoir. Qu'ils en soient, ici, de nouveau remerciés. d'un premier chapitre, car le projet de loi que nous examinons dans un calendrier plus que resserré ne suffira probablement pas à éteindre totalement la crise sociale que nous traversons. Dans nos territoires, nous avons tous entendu les revendications d'une bonne partie de nos concitoyens. Elles sont nombreuses, souvent hétéroclites, parfois contradictoires. On les retrouve maintenant dans les cahiers de doléances ouverts dans certaines mairies : une fois encore, les maires sont Les attentes sont fortes ; comment s'en étonner, alors que tant d'efforts ont été demandés à nos compatriotes depuis 2008 pour surmonter la crise financière et que les effets de la reprise de la croissance peinent à se faire sentir dans leur vie quotidienne On doit comprendre cette envie de bénéficier, enfin, des fruits de tous les efforts qu'ils ont pu consentir. Les signaux ne manquaient évidemment pas, l'exaspération fiscale n'en étant qu'un symptôme paroxystique.

La société dans son ensemble subit ainsi les effets de décisions parfois déconnectées des réalités en point d'en devenir abstraites. Face à une action publique devenue hypertrophiée, illisible, l'urgence sociale, quant à elle, est bien réelle. L'urgence, c'est d'abord de permettre à chacun de vivre dignement, y compris, et surtout, des fruits son travail.

plafonnement, avec les améliorations introduites par nos collègues députés, qui apportent davantage de clarté. Il appartient désormais aux entreprises qui le peuvent de prendre leur part de cet effort collectif. concerne les exonérations de fiscalité et de cotisations sociales des heures supplémentaires et complémentaires, l'accélération du calendrier apportera un gain immédiat de pouvoir d'achat, qui soulagera de nombreux ménages. Le rétablissement du taux de CSG à 6,6 % pour les retraités percevant moins de 2 000 euros nets est également une mesure attendue et de bon sens, qui avait été défendue par une majorité de sénateurs. quel sera, à présent, le calendrier du déploiement de cette mesure ? Enfin, pour ce qui concerne l'article 4, le rapport demandé au Gouvernement doit absolument identifier les moyens de renforcer l'accès de chacun à ses droits, en l'occurrence à la prime d'activité. Après ces quelques considérations circonstanciées, ne soyons pas toutefois naïfs. Pour importantes qu'elles soient, ces avancées demeurent tardives et ne suffisent pas, en elles-mêmes, à répondre à un malaise beaucoup plus profond. Une partie de mes collègues du RDSE continuent de s'interroger sur la réelle universalité des hausses de rémunérations annoncées, y compris celles qui sont liées à la prime d'activité, lesquelles ne relèvent pas- on le sait -de ce texte. De même, l'efficacité de la prime de pouvoir d'achat favorise d'abord les salariés d'entreprises en bonne santé financière. Alors que le besoin de justice sociale est criant, prenons garde à ne pas ajouter de nouvelles frustrations aux colères qui se sont exprimées ces dernières semaines.

et j'ai tendance à dire surtout, en attente d'écoute, d'empathie, d'une autre façon de gouverner garantissant davantage de libertés et d'équité, notamment dans l'accès aux services publics, qu'il s'agisse de l'éducation ou de la santé. Pour paraphraser Marcel Gauchet, il nous faut collectivement réenchanter la démocratie, par l'invention de nouvelles formes d'action publique. Très bien ! À cet égard, le grand débat national voulu par le Président de la République ne doit pas être une nouvelle occasion manquée, d'autant qu'il n'y en aura peut-être pas d'autre Le Sénat tiendra toute sa place dans ce débat, vous l'imaginez bien, tout comme, cela va sans dire, les membres de mon groupe. Aux côtés des autres corps intermédiaires, nous continuerons à être des élus de terrain, à l'écoute des territoires, pour construire collectivement le nouveau contrat social dont notre pays a besoin. a besoin. Comme le disait Nelson Mandela : « Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir.

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, en quelques mois seulement, Emmanuel Macron et son orchestre auront plongé notre pays dans une triple crise, économique, sociale et identitaire, à laquelle est venue s'ajouter la pire de toutes, peut-être, pour le Gouvernement, la crise de confiance. Et pour cause : si vous voulez suivre les agissements, ou plutôt les aventures, de ce qui ressemble de plus en plus à une bande de pieds nickelés, mieux vaut avoir le pied marin ... Chaque jour voit en effet son revirement, son reniement, son renoncement, son rétropédalage, son cafouillage, son changement de cap. Désormais, Édouard Philippe prend moins le chemin de Matignon que celui de Canossa. La Macronie, ce petit bijou de la navigation politique, est devenue en quelques semaines un bateau ivre ! Ce n'est plus le, c'est le- les amoureux de l'oeuvre de Marcel Pagnol me comprendront. L'orthodoxie financière a laissé la place à ce qui ressemble à une fuite en avant. Mais, qu'ils portent un gilet jaune, un uniforme bleu ou une blouse blanche, nos compatriotes ne se laissent plus tromper par les bonimenteurs de l'exécutif, qui accordent du bout des doigts ce qu'ils leur avaient déjà pris, avant de le leur reprendre, et doublement, entre la bûche et le gâteau des rois. Les légitimes revendications salariales des policiers, des enseignants, des agents de la fonction publique hospitalière, en attendant les autres, sont les prémices d'un développement de la crise. Le prélèvement à la source, qui entrera en vigueur au mois de janvier prochain, ne fera que propager l'incendie. Pourtant, de l'argent, il y en a ! À preuve, madame la ministre du travail, voilà à peine deux mois, vous avez su débloquer 15 millions d'euros ! Il s'agissait de les aider à trouver un emploi. Nos compatriotes au chômage apprécieront ce qui ressemble à une véritable provocation

Cette gigantesque fraude coûte la bagatelle de 20 milliards d'euros par an. Voilà un scandale qui mérite assurément la création d'une commission d'enquête parlementaire. Vos économies sont donc toutes trouvées, et elles pourraient permettre de répondre à la souffrance sociale des Français. Mais, au-delà de l'aspect financier, nos compatriotes souhaitent ardemment être écoutés une démocratie réellement représentative. Le Rassemblement national est le seul à proposer, depuis des décennies, l'instauration à la fois du référendum d'initiative populaire ou citoyenne ... Mais il ne veut pas augmenter La restauration d'une confiance fiscale par la suppression des taxes confiscatoires, par des impôts justement répartis, et la restauration de la confiance démocratique par un peuple redevenu souverain rétabliront la confiance de nos compatriotes en la politique. Puisqu'il me reste quelques secondes, je profite de ma présence à la tribune du Sénat pour répondre, de façon symbolique, à la crise identitaire et à la volonté farouche et légitime des Français de défendre leurs traditions et leurs racines, en vous souhaitant, monsieur le président,

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous examinons ce projet de loi dans un contexte préoccupant, qui a vu depuis plusieurs semaines la violence prendre le pas sur le débat démocratique, qui a vu certains irresponsables extrémistes appeler à la disparition de nos institutions républicaines, et qui a vu monter une colère populaire couvant depuis plus de trente à laquelle le gouvernement actuel a sa part de responsabilité, par son manque de dialogue et son obstination difficilement compréhensibles. Votre gouvernement doit reprendre la main pour que notre pays sorte de cette crise par le haut en s'appuyant sur les corps intermédiaires. Comme l'a rappelé Claude Malhuret, c'est au Parlement que l'on fait la loi, et non sur les ronds-points. Eh oui ! Le Sénat, qui a un rôle majeur dans ce pays, a été force de proposition tout au long de la crise, notamment lors de l'examen du projet de loi de finances. Un grand nombre de ses préconisations ont été retenues- un peu tard, il faut le dire -par le Gouvernement. En effet ! Je veux notamment parler du gel de la hausse de la fiscalité énergétique. Quelles sont les causes de la colère ? Quel est le déclencheur ? C'est une vision de l'écologie trop punitive, ... Eh oui ! ... trop peu adaptée aux territoires, trop décalée par rapport à la réalité de ce que vivent nos concitoyens. La voiture n'est pas un ennemi : c'est le gagne-pain de millions de nos concitoyens. Pourquoi prendre les automobilistes pour des vaches à lait ? Je pense au contrôle technique, à la hausse du prix des carburants, à l'heure, dont le Président de la République aurait dit récemment que c'était « une connerie » ! Pourquoi les maintenir, d'autant que les résultats sont loin d'être probants ?

Pour éteindre l'incendie, il fallait revenir sur ces hausses indiscriminées ; le Gouvernement reprend certaines propositions émanant du Sénat- il faut le dire -, et c'est une

malaise d'un travail parfois difficile et pénible, qui ne rapporte pas assez pour permettre de vivre dignement ; malaise, enfin, d'une partie de la population, qui ne se sent plus écoutée par ceux qui dirigent. C'est au Gouvernement de proposer des solutions concrètes, face aux revendications légitimes qui se sont exprimées ces dernières semaines, tout en étant attentif, naturellement, aux propositions du Parlement.

Ce thème est au coeur du présent texte, avec l'exonération d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires.

Ce n'est pas l'idéal, mais c'est une première avancée pour nos concitoyens, et elle mérite d'être notée. L'urgence est également de faire un geste pour les retraités les plus modestes, qui ont été trop taxés par le Gouvernement. Ce projet de loi annule l'augmentation de la CSG subie en 2018 par les retraités dont la pension mensuelle nette était comprise entre 1 400 euros et 2 000 euros. C'est une décision

vous ouvrirez la porte aux extrêmes, avec des conséquences catastrophiques. Prenez garde, le risque est grand ! En démocratie, le pouvoir ne peut ignorer les forces vives de la Nation.

La question est maintenant de savoir si vous parviendrez à aller plus loin que ces mesures de crise pour sortir, enfin, la France de l'ornière. Nous partageons la même préoccupation : ne perdons plus de temps !

au sentiment de relégation d'une partie des Français s'ajoute le rejet du consentement à l'impôt pour former un cocktail explosif. Mes chers collègues, je veux dire un mot de la prime d'activité. Nous sommes favorables à son augmentation, car, dans notre pays, le travail faiblement qualifié paye trop peu.

déjà suffisamment lourd. Le groupe Union Centriste n'oublie pas que la dette d'aujourd'hui se traduit toujours par les impôts de demain. Pour nous, le financement de ces 10 milliards d'euros doit être équilibré par une diminution de la dépense publique et, forcément, par une réforme de l'État.

que la France était prête à renoncer à son histoire sociale et à ce qu'elle considère comme son identité : ses 36 000 communes, ses services publics et son goût pour la justice sociale ; vous avez pensé avoir été élus pour convertir le pays au modèle anglo-saxon, à une organisation libérale du travail dans laquelle la loi s'efface devant le contrat,

vous avez fait le choix d'une politique fiscale anti-redistributive en préférant la à l'ISF. Vous avez cru que les Français allaient tranquillement s'asseoir dans la plaine en attendant que les « premiers de cordée » fassent ruisseler la richesse ! Depuis le 17 novembre, vous découvrez de baisser les impôts des très riches et de libérer la finance tout en augmentant les impôts des autres et en diminuant les dépenses publiques débouche sur une équation insoutenable. collègues étiez tellement obnubilés par votre vision de la modernité, tellement convaincus de la nécessaire mise en conformité de la France au dogme libéral, tellement persuadés que le XXI siècle n'avait commencé que le 7 mai 2017, que vous êtes passés à côté de l'essentiel le besoin de justice sociale et la contestation d'un système économique intrinsèquement injuste, que votre politique fiscale a rendu plus injuste encore. Cette semaine, vous auriez pu corriger cette politique fiscale : le Sénat avait voté à l'unanimité un dispositif contre les montages fiscaux permettant aux titulaires d'actions de mettre leurs portefeuilles à l'abri en les exilant

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est supposé éteindre l'incendie du mouvement social et, surtout, le priver du fort soutien dont il bénéficie dans la population. Prime exceptionnelle à la discrétion des employeurs, défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires, élargissement de la prime d'activité, le tout, sans recettes fiscales nouvelles,

La saison 1 du quinquennat va s'achever ce soir avec le vote de la loi ; personne ne sait encore ce qui va se passer dans la saison 2, mais vous abordez l'année 2019 sous haute surveillance démocratique et sociale. Haute surveillance démocratique, d'abord, car la séquence qui vient de s'achever a considérablement dégradé la parole publique.

trop de com', trop d'amateurisme, trop d'improvisation, sans parler de la mise en scène ridicule d'un bras de fer entre le Président de la République et la technostructure. Quand on connaît le Président de la République et son entourage, cela ne manque pas de sel

se montrer très persuasif pour convaincre que votre réforme n'a pas pour finalité de réduire le montant des pensions. Lever la présomption d'injustice qui pèse désormais sur votre politique ; voilà, mesdames les ministres, votre ordre du jour pour l'année 2019

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, le mouvement des « gilets jaunes » est sans précédent dans la forme : né de la base, répercuté par les réseaux sociaux, il n'a pas fait appel aux organisations qui structurent habituellement la vie sociale de notre pays. Spontané, il a rapidement été massif et distribué sur tout le territoire, principalement, d'ailleurs, en dehors des grandes villes. Ce mouvement social est aussi intéressant et original

elles comptent chaque euro pour nourrir leurs enfants, les habiller dignement et les loger correctement ; elles sont contraintes d'économiser pour le strict nécessaire et ne peuvent se permettre le superflu ; elles culpabilisent de ne pas pouvoir leur offrir une place de cinéma ou une sortie dans un parc d'attractions.

Sans revenir sur les conséquences de cette disposition pour les comptes publics, je tiens à rappeler que toute incitation aux heures supplémentaires est un nouveau frein à l'égalité salariale. En 2015, 56 % des salariés hommes ont eu recours aux heures supplémentaires, contre seulement 38 % des femmes.

en aucun cas, des fraudes. Ces anomalies ne signifient pas qu'il y a eu plusieurs numéros ou que l'assuré n'existe pas. Les cas de fraude au NIR sont rarissimes et je vais donner un exemple qui concerne l'assurance maladie. La délégation nationale à la lutte contre la fraude

les exonérations prévues à l'article 1 ne concernent que les seules primes versées aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le SMIC. L'instauration d'un tel plafond est susceptible de faire naître un effet de seuil.

Pouvant être versée depuis le 11 décembre dernier et jusqu'au 31 mars 2019, cette prime exceptionnelle est source de questionnements pour les plus petites structures, qui, où elles disposent des fonds nécessaires, ne peuvent s'appuyer sur un service des ressources humaines pour lever les doutes concernant son versement et pour la mettre en oeuvre rapidement. Nous voyons fleurir depuis quelques jours un palmarès des entreprises qui jouent le jeu et de celles qui ne se sont pas prononcées.

après plusieurs semaines de mouvements sociaux d'une virulence rarement égalée au cours de ces dernières années, l'exécutif s'est enfin décidé à agir. Sa réponse, préparée dans l'urgence, n'est, hélas ! pas à la hauteur des attentes d'une partie de la population précarisée, légitimement au bord de l'implosion. Les solutions proposées, peu abouties, peu réfléchies et non budgétisées, l'illustrent parfaitement.

La carotte est maigre et l'on porte au passage un énième coup de rabot au financement de la sécurité sociale. Certes, dans le contexte de crise majeure que nous connaissons, je ne peux me résoudre à voter contre une mesure qui pourrait accroître le pouvoir d'achat de certains travailleurs. On peut cependant regretter le caractère non coercitif du dispositif. En laissant l'application de cette mesure au bon vouloir des employeurs, le Gouvernement prend un pari risqué. Au mieux, madame la ministre, vous faites preuve de naïveté en pensant que le patronat fera droit à votre demande. Au pire, vous faites preuve d'insincérité, en promettant beaucoup sans escompter de résultats probants, en misant sur l'essoufflement de la grogne sociale. Soyez sûre que nous serons particulièrement attentifs à la mise en place de cette mesure et que nous tâcherons d'en juger l'efficacité avec rigueur. La

que vous imposez aux plus vulnérables de se serrer la ceinture en ne revalorisant pas les prestations sociales et les pensions de retraite, que les économies demandées entraînent des fermetures d'hôpitaux et de services publics de proximité et portent atteinte à l'accès des

il n'aurait pas les moyens de faire vivre les services publics, mais il a ceux de privilégier les grandes fortunes, puisque le Gouvernement refuse de rétablir l'ISF ! Vous nous répondrez, madame la ministre, que les fonctionnaires sont concernés par le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations

monsieur le président.

d'une salariée en raison de son absence pour congé de maternité n'était ni discriminatoire ni illégale, à condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur l'attribution de cette prime. Cette position a été maintenue le 1 décembre 2016 par la chambre sociale de ladite cour.

et effective de la salariée à certaines activités. Ces décisions sont d'autant plus gênantes qu'elles respectent pleinement les textes et la jurisprudence européens, qui se veulent protecteurs des salariées enceintes ou en congé de maternité. De fait, la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé à plusieurs reprises- et encore le 14 juillet 2016 -qu'une salariée ne pouvait se fonder sur la directive du 19 octobre 1992 assurant la protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes au travail pour revendiquer le maintien de sa rémunération dite « intégrale » pendant son congé de maternité, comme si elle occupait effectivement, comme les autres salariés, son poste de travail. À notre sens, dans ce cas de figure, la salariée est bel et bien victime d'une discrimination indirecte, puisque le congé de maternité est un congé légal obligatoire. Ces décisions sont regrettables et n'envoient pas un signal positif aux femmes, pour lesquelles, bien souvent, le congé de maternité constitue un frein à la carrière professionnelle. Pour toutes ces raisons, nous voulons être certains que les femmes concernées bénéficieront de l'entièreté de la prime et que celle-ci ne leur sera pas versée au prorata du temps passé dans l'entreprise.

de vote sur l'article 1. Nous nous abstiendrons sur l'article 1. Il est certain que la prime sera appréciée comme une augmentation de pouvoir d'achat par celles et ceux qui pourront en bénéficier.

tombe dans les travers de l'« ancien monde » et décide de ressortir du placard une vieille recette libérale déjà utilisée par le passé par Nicolas Sarkozy, celle de la défiscalisation des heures

Destructrice d'emplois, la défiscalisation des heures supplémentaires n'incite nullement les chefs d'entreprise à embaucher de nouveaux salariés. Le bilan est lourd, avec 100 000 emplois perdus pendant le quinquennat de

C'est d'ailleurs pour cette raison que la suppression de ce dispositif avait été mal comprise par les Français lors de la précédente mandature. Au fond, la véritable cause de la crise sociale réside dans le niveau trop faible des rémunérations. La solution trouvée par le Gouvernement semble à cet égard

qui sont le plus incitées à effectuer ces heures supplémentaires défiscalisées, à seule fin de vivre mieux, au détriment parfois de leur santé. Nous prenons acte de l'absence de prise

Supprimer l'impôt et les cotisations sociales peut avoir un effet immédiat et permettre aux salariés d'avoir un peu plus d'argent à la fin du mois. Mais, en réalité, cela les appauvrit considérablement.

rien que pour la sécurité sociale. Or ce sont ces recettes qui financent les services publics de proximité ; ce sont ces recettes qui financent les hôpitaux ; ce sont ces recettes qui permettent le versement d'allocations sociales et de pensions de retraite. En réalité, le peu que les salariés gagneront à la fin du mois, ils le perdront à terme ! De plus, ces mesures de défiscalisation des heures supplémentaires ont un effet néfaste sur l'économie, déjà démontré à plusieurs reprises et dénoncé lors de plusieurs de nos interventions.

libérale à l'oeuvre depuis plusieurs décennies. Sans coûter un centime de plus aux grandes entreprises, elles font reposer sur les salariés la responsabilité de s'assurer un niveau de vie décent en travaillant toujours plus. Or, selon nous, ce sont les employeurs qui se doivent de rémunérer le travail à sa juste valeur.

Pierre Laurent. Nous proposons de procéder à une revalorisation minimale des prestations sociales, à hauteur de l'inflation. Le code de la sécurité sociale prévoit que les prestations sociales doivent faire l'objet d'une revalorisation annuelle visant à prendre en compte l'inflation. Cette revalorisation permet donc sinon d'augmenter le pouvoir d'achat, du moins d'éviter qu'il ne diminue

Les allocations sociales ont pour but de garantir un revenu minimal aux personnes en situation de précarité, qui ont des ressources limitées. Nous considérons que ne pas les revaloriser à hauteur de l'inflation revient à donner un coup de rabot supplémentaire à un système de solidarité déjà bien mal en point. Vous justifiez cette mesure par la nécessité d'assainir les finances publiques. Pourtant, chaque fois que nous faisons des propositions visant à dégager de nouvelles recettes pour l'État, notamment en mettant à contribution les entreprises, les actionnaires et les plus fortunés, vous les rejetez systématiquement.

Nous avons fait le choix d'une revalorisation différenciée et d'efforts spécifiques à destination des Français les plus modestes. Les minima sociaux seront eux revalorisés à hauteur de l'inflation.

de l'aide à la complémentaire santé. Je vous rappelle que nous avons créé une complémentaire santé coûtant moins de 1 euro par jour pour les personnes les plus modestes, celles qui touchent moins de 1 000 euros par mois de pension ou de revenu. Cela représente un gain de 30 euros par mois

Parlementaires communistes, nous sommes opposés au principe même de la CSG, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer à de nombreuses reprises. Je n'y reviendrai pas. Non seulement cette hausse pénalisait les retraités, déjà fort mal traités dans notre pays, mais elle leur faisait aussi payer la légère augmentation du pouvoir d'achat des salariés.

Tant pis pour l'autre moitié ! On n'en est plus à une inégalité près ... Bien sûr, cette disposition sera éphémère et expirera à la fin de l'année 2019, à moins que le Gouvernement n'entende d'ici là les retraités,

parce qu'il apporte tout de même une lueur d'espoir, parce qu'il constitue une petite amélioration pour 5 millions de retraités parmi les plus modestes de notre pays, qui vont attendre le mois de juillet avec impatience. Nous appelons cependant le Gouvernement à étendre son geste à l'ensemble des retraités.

de retirer des moyens à un certain nombre de politiques publiques. Au moment où nous parlons, la pétition « L'affaire du siècle » vient de dépasser le million de signataires, ce qui est considérable.

Nous regrettons que ce que vous appelez des « mesures d'urgence » n'aillent pas jusqu'à la revalorisation des pensions de retraite et des prestations familiales. Je rappellerai l'ensemble des dispositions en faveur de nos aînés que nous avons défendues lors de l'examen du projet de loi de finances,

Nous voterons cet amendement, parce qu'il est juste. Je suis un peu atterrée d'entendre Mme la ministre de la santé essayer de nous démontrer que tout va très bien, madame la marquise, dans le meilleur des mondes, notamment pour les retraités.

et des EHPAD. Ce n'est pas la situation réelle dans le pays ; ce n'est pas la situation de ces établissements ! Je ne doute pas des efforts que vous faites, mais ils sont infinitésimaux par rapport à la situation réelle. Vous accordez de petites choses qui ne correspondent pas à la vie réelle des gens. Vous ne voulez pas entendre, vous persistez et vous signez. La colère

En 2020, les retraités seront donc toujours aussi exposés à la pauvreté ; la hausse de la CSG sera toujours aussi injuste et grèvera toujours autant

parole est à M. Guillaume Gontard. Emmanuel Macron, dans son discours du 10 décembre dernier, a déclaré qu'il voulait que les Françaises et les Français « puissent vivre mieux de leur travail ». Cette volonté, nous la soutenons. C'est pourquoi nous vous présentons cet amendement, dont l'objet est de revaloriser le SMIC à hauteur de 1 760 euros bruts mensuels, à compter du 1 janvier 2020, ce qui correspond à une hausse de 200 euros nets du salaire minimum. Cette revalorisation du SMIC est plus que nécessaire. Les inégalités sociales en France sont de plus en plus fortes, alors que le pays n'a jamais créé autant de richesses. Ces richesses n'ont jamais été aussi mal réparties entre les entreprises et les salariés, entre les « premiers de cordée » et le reste de la population. Nos concitoyennes et nos concitoyens aspirent à plus de justice sociale et refusent de continuer de travailler pour des salaires largement insuffisants. Alors que des millions de personnes sont en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, cette augmentation de 200 euros répond à un besoin fondamental : celui de se loger, de se soigner, de s'alimenter et de se reposer. Je rappelle qu'il faut 1 424 euros nets par mois à une personne seule pour pouvoir vivre décemment, selon un rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il est urgent d'entendre la colère qui s'est exprimée ces dernières semaines, de milliers de citoyennes et de citoyens qui n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois. Cela est d'autant plus vrai pour les femmes, notamment pour celles qui sont seules avec des enfants. Ces femmes sont les plus exposées aux bas salaires, aux emplois précaires et aux temps partiels subis, faut-il encore et toujours le répéter !

Sur le fond, le décret de revalorisation du SMIC a été adopté en conseil des ministres le 19 décembre dernier. Au 1 janvier 2019, le SMIC sera bien augmenté de 1,5 %, conformément aux règles de calcul automatiques prévues par le code du travail.

versé par l'entreprise et d'une forme de solidarité permet l'augmentation des revenus des travailleurs modestes, ce qui est essentiel. La prime

L'entreprise privée et particulièrement les patrons doivent mieux répartir l'argent entre le capital et le travail. Qu'il y ait autant de dividendes distribués et pas assez d'augmentations de salaire, personnellement, ça me choque. Lorsque les Français demandent une augmentation de leur pouvoir d'achat par leur salaire, c'est bien aussi une critique de notre système capitaliste. » Alors, oui, il y a bien un problème de la répartition de la richesse produite par les entreprises

ayant renoncé à la contribution des plus aisés à cet effort en faveur des plus précaires, l'annonce de la revalorisation du SMIC pouvait nous faire craindre le pire, mais il semble avoir évité certains écueils. Le Premier ministre, redoutant de voir sa mesure retoquée par le Conseil constitutionnel, a renoncé à augmenter le salaire minimum net par le biais d'une baisse des cotisations sociales. De même, il pouvait se révéler problématique de faire passer la hausse des bas salaires par la prime d'activité, alors que seuls certains salariés peuvent actuellement en bénéficier, et ce sur demande. En élargissant la base des bénéficiaires de cette prime, en prévoyant l'automaticité de son versement par les CAF et en rendant son recours plus lisible, le Gouvernement semble avoir mis en place un dispositif plus ou moins raisonnable. Bien sûr, nous aurions préféré une augmentation substantielle du salaire brut, à l'image de ce qu'ont récemment fait nos voisins espagnols. Fallait-il encore que l'exécutif ait du courage politique et un véritable temps de réflexion pour entreprendre une telle mesure, sans compter évidemment ses choix antérieurs antérieurs en la matière, qui le bloquent, et auxquels s'ajoute son amateurisme de ces derniers jours ! Le problème majeur que pose en fin de compte cette mesure est son coût 2,5 milliards d'euros, ce n'est pas rien ! Cela aurait pourtant facilement pu être couvert par la réinstauration de l'ISF ou encore une meilleure utilisation du CICE.

au 1 janvier 2019. Je profite de l'examen de cet article pour revenir sur les annonces du Gouvernement. Emmanuel Macron, lors de son discours du 10 décembre dernier, a annoncé que les salariés au SMIC gagneraient 100 euros de plus par mois.

Or il s'agit d'une allocation sociale, versée sous conditions de ressources tenant compte de l'ensemble des revenus du ménage. En raison de ces conditions restrictives, au moins 45 % des salariés au SMIC seraient exclus de cette mesure. Les premières concernées seront évidemment les femmes. De nombreuses femmes recevant de bas salaires n'en bénéficieront pas, parce que leur époux gagne trop. C'est pourquoi nous avions déposé un amendement visant à individualiser le bénéfice de la prime d'activité,

Il me semble qu'il est plus que temps de dépasser cette conception patriarcale et archaïque et d'individualiser les droits, d'autant que les femmes constituent 90 % des personnes recevant

Par ailleurs, cette mesure crée une confusion entre rémunération du travail et solidarité nationale. On demande à cette dernière de compenser les salaires trop faibles versés par les entreprises.

parce qu'il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de technicité et beaucoup de subtilité dans le peuple. Quand on veut bien les écouter, ils nous parlent de justice

Le pouvoir d'achat ne se résume pas au montant net sur sa fiche de paye, à celui de sa pension de retraite ou aux prestations sociales. Les charges incompressibles, au premier rang desquelles le loyer, pèsent lourdement sur les ménages, et proportionnellement plus sur les ménages modestes. Dans notre pays, nous avons la chance d'avoir un système de santé où le reste à charge pour les familles est parmi les plus bas. Nous avons réussi à le réduire encore sous le quinquennat de François Hollande, tout en assainissant les comptes de la sécurité sociale. Ainsi, la part restant à la charge des ménages a continué de reculer, pour s'établir à 7,5 % de la consommation de soins et de biens médicaux en 2017. Cet acquis, nous entendons le conserver, car il garantit un haut niveau de prise en charge à l'ensemble de nos concitoyens. La remise en cause de la compensation intégrale du coût des allégements de charges par l'État et, pire, l'instauration d'une règle inverse, basée sur le principe de non-compensation à l'avenir, sont un très mauvais coup porté à la protection sociale des Français et à leur pouvoir d'achat futur. Car ce gouvernement attend de la part de la sécurité sociale une solidarité financière à l'égard du budget de l'État au moment même où il aggrave le déficit, y compris avec ces mesures dites « d'urgence ». Les excédents attendus de la sécurité sociale doivent rester à la sécurité sociale et servir au

Trop de certitudes, trop d'arrogance, trop d'intelligence ... Vous êtes déconnectés des Français : incompréhension, imprévision et, en cette période, on pourrait même parler d'incompétence. Les Français ont exprimé un besoin de justice, de reconnaissance, de respect. Sans eux, vous continueriez à vous égarer et mèneriez le pays à de grandes difficultés, fragilisant fondamentalement notre modèle social. Je me souviens des éléments de langage des ministres : « Macron ou le chaos ». Dans les faits, nous avons eu Macron et le chaos. Exactement ministres, votre mouvement venu de nulle part a été submergé par un mouvement venu de partout ; je ne fais que citer notre collègue Pierre Ouzoulias. Les mesures que vous nous proposez sont insuffisantes pour les fonctionnaires, pour les retraités

locales ; des CCAS seront en grande difficulté pour faire face à leurs obligations sociales. Votre financement est déséquilibré. Il repose trop sur la solidarité nationale et pas assez sur

C'est totalement faux ! En 2012, 587 redevables de l'ISF avaient quitté le territoire, soit un nombre faible et stable, d'après la direction générale des finances publiques, pour un manque à gagner de 270 millions d'euros pour l'État.

le mouvement des « gilets jaunes » est un cri de colère, mais aussi un cri existentiel. On ne peut pas réduire ses revendications aux seuls aspects matériels. Il y a un sentiment de relégation, relégation, sans doute sociale et économique, mais également territoriale et civique. M. le président de la commission des affaires sociales a parlé d'« abaissement ». Oui, il y a un sentiment d'abaissement ! Il faudra bien autre chose pour que le problème puisse être réglé au fond.

on ne souffle pas sur les braises encore rougeoyantes de la colère. C'est une évidence ! D'autre part, au moment où c'est la légitimité qui est atteinte, pas seulement celle du

très rapidement dans ce projet de loi. La procédure est évidemment exceptionnelle par sa brièveté ; elle l'est aussi par son ampleur, comme cela a été souligné sur différentes travées. Il fallait sans doute éteindre l'incendie et donner des signaux de compréhension de la colère qui s'est exprimée et des difficultés du déclassement vécues par les classes moyennes dans notre pays. Nous avions été nombreux dans cet hémicycle à alerter sur la désindexation des retraites, sur la CSG pour les retraités et sur d'autres mesures qui n'ont pas été comprises et qui, traduites d'une manière pour le moins imparfaite, ont été à la source d'une partie des difficultés. Le Sénat a abordé la discussion dans un esprit de responsabilité. Nous nous sommes centrés sur l'obligation de sortir par le haut d'une crise exceptionnelle qui ne peut pas durer.

Les solutions d'urgence ne sont jamais parfaitement satisfaisantes. Elles sont là pour répondre à une situation grave, à un moment donné. On ne pouvait évidemment pas balayer d'un revers de main le mouvement des « gilets jaunes », qui traduit véritablement un profond malaise.